La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification,

une mission sur l’évolution du travail parlementaire, en ma qualité de présidente de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire et des conditions d’exercice du mandat de sénateur. Cette mission m’a amenée à entendre l’ensemble des présidents de commission, de délégation et de groupe, mais aussi des personnalités extérieures, parmi lesquelles plusieurs de nos collègues du parlement italien. De ces échanges fructueux sont ressorties dix sept propositions, qui ont été adoptées par la conférence des présidents et qui peuvent être réparties selon quatre axes : conforter notre procédure législative pour renforcer le rôle du Parlement tout en préservant la qualité du débat parlementaire renforcer nos moyens de contrôle ; simplifier la gestion de l’agenda de nos collègues ; enfin, poursuivre l’adaptation de notre règlement aux évolutions de nos pratiques. Plusieurs de ces 17 propositions sont déjà mises en œuvre par la conférence des présidents. C’est le cas de la nouvelle organisation de nos mardis après midi des semaines de contrôle, qui sont désormais consacrés aux travaux des délégations, des structures temporaires et des commissions. Il s’agit à la fois de renforcer le contrôle – vous êtes nombreux à estimer qu’il est plus efficace en commission et devant les délégations –, mais aussi de permettre à un plus grand nombre de nos collègues d’assister aux différentes réunions qui, jusqu’à présent, avaient tendance à se chevaucher. C’est également le cas de la réorganisation de nos semaines sénatoriales : l’espace réservé du mercredi après midi de la semaine d’initiative a été déplacé au mercredi de la semaine de contrôle, afin, d’une part,

Le premier espace a été mis en place le mercredi 19 mars dernier, avec l’examen de deux propositions de loi et d’une proposition de résolution, en application de l’article 34 1 de la Constitution, toutes trois adoptées à l’unanimité. Il s’agit là d’une occasion de valoriser et de faire prospérer les initiatives parlementaires faisant l’objet d’un large consensus au sein de notre assemblée, un esprit de coconstruction et de travail en bonne intelligence entre les différents groupes. Le second espace transpartisan aura lieu le mercredi 14 mai prochain et connaîtra, je l’espère, le même engouement.

Ces mesures visent, par exemple, à reconnaître un intérêt à agir aux présidents des commissions et des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat en matière d’application des lois, ou encore à enrichir les dispositions relatives aux études d’impact et à soumettre les amendements du Gouvernement à une obligation de production d’étude d’impact. Elles devront être adoptées par l’Assemblée nationale pour pouvoir être mises en œuvre. J’en viens maintenant aux mesures qui modifient notre règlement et qui sont soumises à votre approbation ce soir. Plusieurs d’entre elles visent à conforter les droits des groupes politiques. Tel est le sens de l’article 2, qui attribue aux groupes la « propriété » de leurs postes au sein du Bureau, ainsi que des commissions et des structures temporaires. En cas de changement de groupe, le sénateur concerné cesserait de plein droit d’appartenir à cette instance. Le groupe « propriétaire » du poste aurait le choix de nommer un sénateur à sa place ou de laisser le poste. Il s’agit là d’une demande forte qui a été exprimée par l’ensemble des groupes de notre assemblée. Il appartiendra au Bureau d’édicter cette même règle pour les présidences et pour le bureau des groupes d’études et des groupes d’amitié. Plusieurs mesures portent par ailleurs sur le renforcement des missions de contrôle et s’inscrivent dans la continuité des conclusions de la mission de réflexion sur le contrôle sénatorial, dont notre collègue Pascale Gruny, alors vice présidente du Sénat, était le rapporteur. Ainsi, l’article 7 simplifie l’octroi des prérogatives de commission d’enquête aux commissions permanentes, en remplaçant le passage en séance publique par une procédure d’affichage et de ratification en l’absence d’opposition. L’article 19 réécrit le chapitre XX du règlement, relatif aux affaires européennes. Il est notamment proposé de clarifier la rédaction actuelle en distinguant mieux la procédure à suivre, selon qu’une proposition de résolution européenne est engagée par la commission permanente, par la commission des affaires européennes ou par un sénateur. En outre, les propositions de résolutions européennes déposées par les sénateurs ne seraient plus automatiquement examinées par la commission des affaires européennes, mais pourraient l’être à la demande d’un président de groupe ou de commission. En complément, j’ai proposé qu’un vade mecum vienne préciser les bonnes pratiques d’élaboration des propositions de résolution déposées au nom de la commission des affaires européennes, notamment le délai de mise à disposition du projet de texte du rapporteur aux autres membres de la commission, afin de leur permettre de proposer des amendements. Ce vade mecum pourrait également œuvrer dans le sens d’un renforcement des interactions entre la commission des affaires européennes et les commissions permanentes, en prévoyant une veille active alertant les sénateurs des initiatives législatives européennes susceptibles d’affecter le droit national. Par ailleurs, la proposition de résolution comporte diverses dispositions destinées à sécuriser notre règlement. Par exemple, l’article 21 modifie l’article 96 du règlement, afin de de renforcer le caractère collégial et contradictoire de la procédure de sanction en matière de censure : il transfère le pouvoir de proposition de cette sanction, qui emporte des conséquences financières importantes, du président du Sénat au Bureau. Il s’agit ici de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui exige que le parlementaire sanctionné bénéficie de garanties procédurales. Dans le même esprit, la présente proposition de résolution prévoit des mesures d’actualisation du règlement, pour le rendre plus conforme aux pratiques. Je citerai notamment l’article 11, qui procède à une actualisation du rôle des secrétaires en cas de scrutin public ordinaire, pour tenir compte de la mise en place du système de scrutin électronique.

Enfin, plusieurs articles de la présente proposition de résolution suppriment des mesures obsolètes du règlement et corrigent des erreurs de coordination. Ainsi, l’article 22 abroge l’article 106 du règlement relatif aux députations, qui permettait d’envoyer dans les cérémonies une députation, c’est à dire des membres de l’assemblée concernée tirés au sort. Cette disposition n’ayant jamais été utilisée depuis 1959, je vous propose de la supprimer. La réflexion doit encore se poursuivre sur les outils qui pourraient nous être utiles demain si le développement de l’intelligence artificielle et un recours accru à cette technologie entraînaient une démultiplication du nombre d’amendements et si les outils du règlement du Sénat apparaissaient insuffisants pour y faire face. Mes chers collègues, je vous rappelle l’exemple du Sénat italien, où un vice président a déposé 83 millions d’amendements… Aujourd’hui, seul le Gouvernement peut agir face à une telle situation, avec les outils que la Constitution lui a confiés. Cela crée un biais qu’il nous faut résoudre : le Sénat doit pouvoir anticiper les grandes évolutions, mais aussi réagir rapidement aux enjeux plus immédiats. Il y va de notre responsabilité individuelle et collective, par delà nos sensibilités distinctes. En conclusion, je suis convaincue que ces mesures, qui ont été élaborées en tenant compte des observations qui m’ont été faites, sauront recueillir un consensus autour d’un objectif qui doit tous nous rassembler : l’amélioration des conditions du travail parlementaire. Plus que jamais, le Sénat doit continuer d’incarner une assemblée efficace au service de tous nos concitoyens, qui ne transige jamais sur la qualité du débat et veille au respect de nos différences, tout en sachant transcender les clivages au nom de l’intérêt général. Je remercie Mme le rapporteur de l’examen attentif et pertinent du texte Je remercie bien sûr, et sans réserve, l’équipe de la séance et le cabinet du président Larcher, qui m’ont accompagnée avec patience et bonne humeur depuis plus d’un an et qui méritent eux aussi votre soutien. La parole est à Mme le

Madame la présidente, mes chers collègues, cette proposition de résolution fait suite aux travaux, placés sous l’égide du président Larcher, de notre collègue Sylvie Vermeillet, vice présidente du Sénat, dans le cadre de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire et des conditions d’exercice du mandat de sénateur. Ces travaux visent principalement à renforcer le rôle du Parlement dans la procédure législative et à accroître les outils de contrôle des sénateurs. Ils s’inscrivent dans la poursuite de l’adaptation du règlement aux pratiques du fonctionnement de notre Haute Assemblée. Ainsi, 17 propositions ont été adoptées en conférence des présidents.

Je me limiterai ici, dans le cadre du débat qui nous réunit, à évoquer quelques enjeux pour le Sénat. Il convient en effet d’accroître nos moyens d’investigation et de travail, aussi bien ceux du Sénat et de ses commissions que ceux de chaque sénateur, afin que nous puissions mieux légiférer, sans dépendre du Gouvernement. Nous manquons, en dépit de la grande qualité des services du Sénat, de moyens propres suffisants pour mesurer l’impact de telle ou telle proposition. Par ailleurs, l’article 20 de la présente proposition de résolution me fait réagir sur la trajectoire de transparence et de contrôle de la vie politique et des élus dans laquelle nous sommes engagés et qui me semble très préoccupante. Même l’ancien député René Dosière, qui s’est fait connaître comme le Monsieur Propre de l’utilisation de l’argent public, s’inquiétait de ce climat déclarait : « Je suis très inquiet de la manière dont se passent les choses. La transparence, c’est un moyen de mieux faire fonctionner la démocratie quand il s’agit d’argent public. Mais la transparence sur la vie privée, c’est un régime dictatorial, ou moralisateur, enfin c’est l’enfer !

elle est fort heureusement largement répandue. Mais attention à l’effet de balancier, qui risque de dissuader beaucoup de nos concitoyens de s’investir dans la vie publique et qui jette toujours plus la suspicion, pour ne pas dire le soupçon, voire peut être désormais un de culpabilité, sur ceux qui s’engagent.

Quand va t on s’apercevoir que faire de la politique, c’est se mettre à nu et dévoiler sa situation personnelle, laquelle ne relève en rien de l’engagement public ? C’est mettre en difficulté ses proches, leur créer des contraintes supplémentaires. C’est exposer sa vie d’avant et hypothéquer sa vie d’après.

Cette démarche s’est appuyée sur une concertation approfondie avec l’ensemble des présidents de groupe, de commission et de délégation, selon une méthode respectueuse de nos équilibres. Cela mérite d’être souligné. Issue de cette réflexion collective, cette proposition de résolution n’est pas qu’une simple révision technique de notre règlement. Son examen intervient à un moment qui est loin d’être anodin : le Sénat se doit d’être pleinement conscient de son rôle dans l’espace démocratique. Dans un contexte où le politique est mis en cause, où la confiance se délite, où la parole publique est attendue au tournant, nous devons plus que jamais nous montrer à la hauteur de nos missions.

Il est communément admis que les débats sont souvent plus apaisés dans cette chambre, qu’il est possible d’aboutir à des compromis et, plus largement, que l’examen des textes a lieu avec une certaine sérénité. Cette capacité à nous extraire des logiques partisanes constitue notre force. Elle fonde la légitimité de notre rôle de contrôle, un rôle que nous devons pleinement assumer. Cette proposition de résolution répond clairement Elle renforce les prérogatives des commissions, facilite l’octroi des pouvoirs d’enquête, introduit des créneaux de contrôle plus lisibles et permet d’auditionner à mi parcours les personnalités nommées au titre de l’article 13 de la Constitution. Ces outils ne sont pas de simples accessoires institutionnels : ils traduisent une exigence de transparence, de rigueur et d’évaluation qui est au cœur d’une démocratie vivante. Le texte va plus loin : il conforte les droits des groupes politiques, en reconnaissant leur rôle structurant dans la répartition des responsabilités, et clarifie des points essentiels pour éviter que nos règles ne deviennent un frein à l’efficacité du travail parlementaire. Il modernise, simplifie, sécurise et supprime ce qui est devenu obsolète. Dans un État de droit, le Parlement n’est pas un spectateur. Il est un acteur, un garant, parfois un garde fou. Quand les équilibres institutionnels sont fragiles, comme c’est le cas de nos devient central. Ce texte, par les outils qu’il met à notre disposition, nous permettra, s’il est adopté, de jouer ce rôle avec plus de force, plus de clarté et plus de responsabilité. Si, à première vue, il semble relever de l’entre soi et n’intéresser que les seuls sénateurs, il sert en réalité l’intérêt de tous. Il tend en effet à renforcer la démocratie, en permettant au Sénat de mieux remplir ses fonctions de contrôle et de représentation et, en définitive, de mieux servir nos concitoyens.

Voilà une bonne mesure, sous réserve que le principe de la répartition des postes à la représentation proportionnelle soit bien respecté. En effet, le droit de « propriété » ne vaut que tant que les effectifs des groupes n’évoluent pas de façon substantielle durant le triennat.

lors de la conférence des présidents du 19 mars dernier, deux textes ont bénéficié du délai normal de deux semaines, tandis que dix huit autres ont fait l’objet de la dérogation l’exception est devenue la règle, au détriment d’un examen serein des textes de loi. La lecture des conclusions des commissions mixtes paritaires (CMP) intervient également trop souvent dans un délai contraint, parfois le lendemain de la réunion.

n’est pas synonyme de précipitation. Au fond, le débat que nous avons aujourd’hui soulève une question plus fondamentale : ne faudrait il pas réfléchir à de nouveaux ajustements constitutionnels ? Un constat s’impose en effet : depuis quelques années et à son corps défendant, la machine parlementaire s’est emballée ; elle tourne à plein régime, de jour comme de nuit […] Mais, chacun a pu le constater,

cent textes en cent jours : tel est, selon le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, le beau bilan de l’activité du Parlement. Je ne sais pas si nous devons nous féliciter de ce qu’il convient plutôt d’appeler une suractivité parlementaire, mais, en tout cas, cela suffit à me convaincre que l’amendement tendant à supprimer les votes par scrutin public par groupe n’est pas bienvenu. Bien entendu, nos votes doivent rester personnels et il nous revient d’être particulièrement vigilants dans les consignes de vote que nous transmettons à nos groupes. il est illusoire de croire que nous pouvons, avec les moyens insuffisants qui sont les nôtres, prendre une part active ou même éclairée à l’ensemble des travaux parlementaires. Nous ne pouvons pas et même nous ne devons pas être partout.

je tiens à le souligner. Il en va ainsi de la clarification de la procédure par laquelle une commission permanente peut déposer une proposition de résolution européenne. Les commissions permanentes pourront se saisir au fond, ce qui, là encore, me semble très intéressant pour améliorer notre connaissance des sujets européens.

De nombreux amendements ont été déposés sur ce texte. Leur examen nous permettra de mener d’intéressants débats. Même s’ils ne devaient pas être adoptés, ils nourriront notre réflexion dans la perspective de prochaines évolutions de notre règlement, que notre président souhaite régulièrement actualiser.

Nous nous honorons de parvenir à des consensus lorsque c’est possible – l’espace transpartisan en est une bonne illustration. Lorsque ce n’est pas possible, la qualité de nos échanges, emprunts de respect, est montrée en exemple. On voit sur certains sujets d’autres majorités se former, et cela participe de la vitalité de nos travaux. Gardons à l’esprit que la majorité d’aujourd’hui peut devenir la minorité de demain. Alors que nous procédons à une modernisation du règlement du Sénat, je vous soumets, mes chers

Nos élus, les conseillers des Français de l’étranger, font un travail de terrain, et nous les accompagnons de notre mieux à distance. Mais rien, nous le savons, ne saurait remplacer les déplacements. Ils ont besoin de notre présence, et nous avons besoin d’aller au contact de leurs réalités, qui sont très diverses.

La légitimité du Sénat repose notamment sur les compétences de ses membres. Ne négligeons donc aucune modalité de travail qui nous permettrait d’en gagner, en utilisant, plutôt que d’en créer, les structures existantes. Ce texte est l’aboutissement d’un travail important, dans tous les sens du terme, et je tiens à réitérer mes félicitations à notre collègue Sylvie Vermeillet. Le groupe Union Centriste votera ce texte. La parole

car ce document garantit le fonctionnement démocratique de notre institution. L’ambition première de cette réforme nous avait inquiétés, car, une nouvelle fois, la majorité de notre assemblée affichait une volonté forte de rationalisation du travail parlementaire, c’est à dire, en langage décodé,

une prise en compte, presque inédite, des remarques émises par les différents groupes – c’est un facteur positif que nous saluons – et, d’autre part, une évolution de la situation politique, qui confère au Parlement une responsabilité nouvelle. Le président du Sénat le sait bien, à chaque réforme du règlement, notre groupe souligne l’incongruité que représente le fait, pour une assemblée parlementaire, de voter elle même la réduction de ses prérogatives, ce qui favorise ainsi le pouvoir exécutif. D’année en année, déposer un amendement est devenu un exercice difficile. D’année en année, développer une argumentation construite est devenu une gageure, tant le temps de parole est restreint. Sur ce dernier point, nous avons souvent alerté sur le fait que la restriction des discussions pouvait paradoxalement alimenter le dépôt d’amendements.

plus fortement encore qu’en juin 2022. La configuration nouvelle place, de fait, le Parlement au centre du jeu, même si, comme François Bayrou l’a confirmé sans ambages, la tentation de le contourner est grande. La recherche de majorités texte par texte exige un débat approfondi et l’expression précise de chaque groupe. Le rôle important, voire décisif, du Sénat dans l’adoption des textes exige également que nous ayons ici, au Palais du Luxembourg, J’ai relevé ainsi, avec un certain étonnement, que l’on voulait réduire les possibilités d’expression contre les conclusions d’une commission mixte paritaire, en écartant, par exemple, la possibilité de déposer une question préalable à leur encontre.

sur le travail effectué par les quatorze parlementaires qui légifèrent dans des conditions de transparence bien modestes. Dans ce contexte éruptif, il était donc difficile de corseter plus encore le travail parlementaire. La démocratie est en crise et il faudra se pencher, dans de proches délais, sur notre Constitution. Le mouvement d’hyperprésidentialisation, accéléré par Emmanuel Macron, a causé des dégâts considérables sur le plan institutionnel et sur la confiance du peuple dans notre système politique.

car c’est dans les articles du texte qui régit nos travaux que se trouvent, selon nous, les clés d’une restauration des prérogatives parlementaires. Nous proposerons donc quelques amendements – bien loin des millions déposés au Parlement italien…

j’ai pu apprécier la qualité des échanges que nous avons lors de nos différents travaux, en partie grâce aux règles qui régissent le fonctionnement de notre institution. J’ai pu aussi, durant ce court laps de temps, observer certaines problématiques liées notamment à l’appartenance à un groupe d’opposition.

Mon groupe accueille très favorablement l’article 20 sur le renforcement des obligations déontologiques. Celles ci pourraient être accrues : je pense notamment aux obligations déclaratives relatives aux voyages offerts par des groupes d’intérêt public ou des États étrangers.

Hormis quelques précisions rédactionnelles bienvenues, mais secondaires, cette réécriture aurait pu et dû mettre en avant le rôle de la commission des affaires européennes, qui n’a cessé de croître au fil des années à mesure que les enjeux européens Pourtant, la réécriture proposée, à force de détails et de répétitions, aboutira à rendre les procédures plus complexes, alors que le règlement actuel nous semble explicite.

Cette commission a su s’imposer au fil des années, par la qualité de son travail et par sa crédibilité. Cette instance est écoutée, aussi bien au sein du Sénat qu’au niveau européen. Elle constitue un atout que nous devons préserver, mais aussi, je crois, renforcer, parce qu’elle est indispensable.

! Si seuls demeurent les écrits, il nous semble nécessaire, sans faire de procès d’intention, que cette évolution démocratique soit enfin inscrite « en dur » dans notre règlement, comme c’est le cas à l’Assemblée nationale.

que d’hommes à ces fonctions. Et si la désignation est en nombre impair, alors l’écart ne doit pas être de plus d’un. Nous devrions pouvoir y survivre collectivement. De même, nous voudrions une parité dans les présidences de commission. Je souhaite évoquer un dernier point : le vote par assis et levé. Cette modalité de vote, qui pouvait apparaître comme une stigmatisation des personnes à mobilité réduite, a été abolie

La pratique sénatoriale du scrutin public constitue une dernière et importante anomalie : elle autorise un unique sénateur à voter pour l’ensemble des membres de son groupe. Cette modalité de vote de vote est de toute évidence contraire à l’article 27 de la Constitution, qui dispose : « Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. » Il nous semble essentiel de revenir à la stricte application de ce texte, comme le font déjà nos collègues de l’Assemblée nationale. Absolument ! Non ! Enfin, nous souhaitons instaurer une règle de révision du crédit dédié aux collaborateurs. Avec la fin des majorités absolues à l’Assemblée nationale, notre chambre a retrouvé une place centrale dans nos institutions. Cependant, nos équipes sont notoirement trop peu nombreuses pour faire face à celles de l’exécutif et leurs rémunérations bien trop contraintes, alors même que notre besoin d’expertise s’intensifie. s’intensifie. Il paraît donc indispensable que l’enveloppe des crédits affectés à la rémunération des collaborateurs soit indexée sur l’inflation. Pour conclure, je confirme que nous adhérons globalement à la philosophie de ce texte. Cette mise à jour est nécessaire, mais nous souhaitons mettre l’accent sur des sujets qui nous paraissent essentiels dans un parlement moderne : les droits de l’opposition, la parité, l’égalité et la transparence.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, c’est un honneur, en tant que délégué de la réunion administrative des sénateurs n’appartenant à aucun groupe (Rasnag), d’évoquer avec vous les règles qui régissent notre institution. Notre règlement est bien plus qu’un simple recueil de procédures : il est la colonne vertébrale de notre travail législatif, et sa modification doit être faite avec parcimonie et mesure. À ce titre, il me faut saluer le travail de concertation parfaitement œcuménique mené par la vice présidente Sylvie Vermeillet. Vous le savez comme moi, nous ne sommes plus seulement dans une crise de confiance : nous faisons face à une défiance généralisée, profonde et installée de nos concitoyens à l’encontre du Parlement, des politiques et de la politique en général. Le règlement du Sénat, loin d’être une simple formalité technique ou procédurale, doit conforter tant l’efficacité de notre travail législatif que les droits des législateurs, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition. Ainsi, à l’instar de nos collègues, nous saluons l’évolution bienvenue de l’article 2, avec la clarification apportée à la notion de « propriété » politique des sièges dans les commissions du Sénat. Cette mesure peut, sur le papier, apparaître comme une réponse logique à certaines pratiques parfois ambiguës. Pour le reste, je sais que l’un des principaux enjeux de cette réforme du règlement était de tenter de fluidifier les débats et de rationaliser le temps en hémicycle. J’imagine que personne n’oserait dire que nous travaillons trop : aucun de nos compatriotes ne le comprendrait, et à raison… Simplement, il a pu arriver que les débats s’éternisent de manière artificielle, en particulier à l’occasion des projets de loi de finances, que ce soit en 2023 ou en 2024. Ce temps, nous devrions parfois le passer sur le terrain, aux côtés des élus locaux et de nos concitoyens ; c’est aussi notre mission, au delà du simple travail législatif. Le véritable problème se situe ailleurs, et j’ai déjà pu m’en ouvrir auprès de vous, mes chers collègues : la réponse n’est pas réglementaire. Elle relève plutôt de la discipline individuelle et collective. La place de plus en plus importante qu’ont prise les réseaux sociaux dans le suivi de la vie politique a modifié nos pratiques, parfois en bien, puisqu’elle démocratise l’accès à l’information, mais souvent en mal, puisqu’elle fait la part belle aux égos et à la tentation de multiplier le nombre d’amendements pour faire des vidéos et remplir les profils Facebook et Twitter. Un parlementaire me confiait que, entre 2005 et 2025, le nombre d’amendements sur les projets de loi de finances avait été multiplié par dix. Nous connaissons également l’autre cause de cette inflation : l’absence de majorité à l’Assemblée nationale fait de notre chambre une institution désormais centrale dans le travail législatif et nous avons tendance à rejouer les matchs. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais nous devons aussi regarder en face les dérives que cette situation peut entraîner. Je ne jette évidemment la pierre à personne, puisque nous cédons tous, à des degrés divers, à de mauvaises pratiques, mais nous voyons bien que l’inflation législative n’est pas toujours utile ni désintéressée. Ce sont des choses sur lesquelles, malheureusement, aucun règlement intérieur ou aucun projet de résolution n’aura de prise réelle. Pour autant, nous n’avons aucune raison de nous opposer à ce texte, qui préserve de manière bienvenue les droits de la Rasnag. Nous le voterons donc. La parole

Madame la présidente, madame le rapporteur, mes chers collègues, dans le contexte politique troublé que notre pays connaît actuellement, le rôle du Parlement, singulièrement celui du Sénat, revient au premier plan. Pour mener à bien ses missions, le Sénat doit veiller en permanence à l’efficacité des dispositions de son règlement. La proposition que nous examinons aujourd’hui vise à adapter nos règles de fonctionnement aux exigences contemporaines de l’action parlementaire, dans un esprit de continuité, d’efficacité et de responsabilité. Fruit d’un travail mené, sur l’initiative du président du Sénat, Gérard Larcher,

Nous avons apprécié l’écoute accordée aux contributions de l’ensemble des présidents de groupe, de commission et de délégation. Le texte qui nous est soumis contient des dispositions techniques, parfois complexes, qui visent toutes à permettre à notre assemblée de mieux exercer ses missions, dans un environnement institutionnel et politique en constante mutation. Afin de renforcer nos outils de contrôle, il est prévu de simplifier la procédure conférant à une commission permanente les pouvoirs d’une commission d’enquête, ou encore de fluidifier la désignation des membres des commissions mixtes paritaires. La procédure d’examen des propositions de résolution européennes (PPRE) fait l’objet d’un article important. Les trois régimes prévus en fonction de la catégorie à laquelle appartient l’auteur de cette PPRE apporteront davantage de clarté, de souplesse et d’efficacité. Il nous semble que ces dispositions sont pragmatiques concourront utilement à la qualité du débat parlementaire. Une attention particulière a également été portée aux droits des groupes politiques. Le texte clarifie notamment l’attribution des sièges dans les organes du Sénat, en assurant une meilleure lisibilité lors des changements d’appartenance politique. De telles dispositions contribueront également à garantir une représentation plus fidèle des équilibres internes. Par ailleurs, plusieurs articles visent à améliorer la lisibilité et la cohérence de notre règlement. C’est notamment le cas des ajustements liés à l’évolution des outils de vote, ou encore d’une révision des modalités de prise de parole en séance.

Comme il est déjà précisé dans le code de conduite, les sénateurs ne peuvent accepter un cadeau offert par un représentant d’intérêts lorsque sa valeur est supérieure à 150 euros.

Cela participe pleinement à l’objectif de simplification. En définitive, cette proposition ne constitue ni une rupture ni une simple mise à jour à jour formelle. Elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue au service de notre institution. Conscient de ses responsabilités et soucieux de son image, le Sénat se donne ainsi les moyens de renforcer son efficacité.

Madame la présidente, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous débattons ce soir d’une proposition de résolution qui vise à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, à conforter les droits des groupes politiques et à introduire diverses mesures de clarification et de simplification du règlement du Sénat. Ce texte s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’amélioration continue de notre institution, en vue de rendre nos travaux législatifs plus efficaces, plus transparents et mieux adaptés aux enjeux contemporains. Je tiens à saluer tout particulièrement le travail effectué par la sénatrice Muriel Jourda, rapporteur de cette proposition de résolution, qui a su, avec diligence et rigueur, mettre en lumière les réformes nécessaires. L’une des mesures les plus marquantes est la simplification de la procédure d’élection du président du Sénat en cas de vacance de cette fonction. En évitant de repasser par le bureau d’âge, cette réforme nous permettra de gagner en rapidité, tout en préservant la rigueur de nos processus. Cette simplification, loin de dénaturer la procédure, vise au contraire à la rendre plus fluide et mieux adaptée aux réalités du terrain. Ensuite, la centralisation de la recevabilité des propositions de commission d’enquête au sein de la commission des lois mérite d’être saluée. En confiant explicitement cette compétence à celle ci, nous assurons une meilleure transparence et une plus grande cohérence de la gestion des demandes. Ce renforcement du contrôle parlementaire est un progrès tangible pour notre institution. La réforme du renouvellement des commissions spéciales est également un élément essentiel de ce texte. Elle introduit une souplesse bienvenue dans notre organisation interne. Jusqu’à présent, les commissions spéciales se reconstituaient de plein droit après chaque renouvellement du Sénat. Désormais, nous n’aurons besoin que d’une validation par la conférence des présidents. La simplification des nominations des membres des commissions mixtes paritaires (CMP) est un autre point important de cette proposition. Actuellement, la procédure de nomination peut sembler trop complexe et lourde. En confiant cette tâche au seul président de la commission compétente, nous simplifierons ce processus, permettant ainsi un gain de temps et d’efficacité. telle mesure s’inscrit dans une logique d’adaptation du règlement à nos pratiques actuelles, pour mieux répondre aux exigences du travail parlementaire. En matière de déontologie, la proposition fait également des avancées notables. En clarifiant les règles concernant les cadeaux et les déplacements offerts aux sénateurs, elle renforce la transparence et la confiance que nos concitoyens doivent avoir en nous. La réécriture des dispositions concernant la commission des affaires européennes est à mes yeux importante. Cette réforme vise à rendre plus fluide l’examen des propositions de résolution européennes, en permettant un traitement conjoint avec la commission compétente sur le fond. Cela renforce non seulement l’efficacité de notre travail, mais aussi notre capacité à répondre aux enjeux européens, qui sont de plus en plus complexes. visant à confier au Bureau, et non plus uniquement au président du Sénat, la responsabilité de proposer des sanctions en cas de dérive d’un sénateur est un gage de collégialité et de transparence dans le fonctionnement de notre institution.

nous le savons, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, si les progrès ne sont pas garantis par les textes, les régressions sont toujours possibles. Il s’agit donc de cranter ce principe dans notre règlement. Quel

est à Mme Maryse Carrère. Les changements du paysage politique et l’abaissement du seuil d’effectif ont conduit à multiplier les groupes politiques au Sénat. Nous avions cinq groupes en 2008, six en 2014 et 2011, sept en 2017 et huit depuis 2020.

Contrairement à l’Assemblée nationale, où les réunions de commission sont retransmises en direct et accessibles en différé, les réunions de commissions du Sénat ne bénéficient pas de telles diffusions. Par conséquent, lorsqu’un sénateur ultramarin ne peut

aux réunions de leurs commissions en visioconférence. Cette mesure vise à améliorer leur accès aux travaux préparatoires des textes de loi et à mieux prendre en compte les contraintes spécifiques qui Nous prévoyons néanmoins deux limites strictes : les sénateurs participant par visioconférence ne pourraient pas voter sur les textes examinés en commission et leur participation à distance ne serait pas assimilée à une présence effective.

Au Sénat, les auditions des rapporteurs renforcent les connaissances du Parlement sur les sujets dont il se saisit et permettent de légiférer en connaissance de cause. Nos collaborateurs en sont pourtant exclus.

Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d’un projet ou d’une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des Présidents, la commission saisie au fond se réunit. » Pourtant, nous constatons tous que l’exception est devenue la règle

les textes et d’exercer leur droit d’amendement dans de meilleures conditions.

il n’y a aucune obligation d’explication des décisions d’irrecevabilité. Le périmètre indicatif, diffusé en amont d’un examen, n’apporte pas l’éclairage suffisant pour comprendre les choix qui ont conduit

collectivement à de nouvelles règles pour une meilleure acceptabilité des irrecevabilités, qui sont nécessaires au bon déroulement de nos débats législatifs.

dans le calcul. À votre bon cœur

Michel Masset. La laïcité est une valeur à laquelle le RDSE, ancien grand groupe du Sénat, est attaché. Inscrite dans notre Constitution, elle est au fondement de notre régime républicain. Dans la vie civile, on observe de plus en plus d’atteintes à la laïcité. Le Parlement doit rester à l’abri de cette dérive. Aussi notre règlement doit il être plus ferme, afin que les sénateurs respectent scrupuleusement

la nouvelle procédure prévoit d’attendre la prochaine réunion du Bureau. Ainsi une contestation pourrait elle rester en suspens pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D’autre part, la nouvelle procédure laisse au Bureau la faculté de refuser

ne peuvent être présents en séance. Cependant, ces dérogations ne couvrent pas les sénateurs chargés par le Gouvernement d’une mission temporaire. Or ces missions, qui leur sont confiées par décret, s’inscrivent pleinement dans le travail parlementaire et contribuent à l’élaboration des politiques publiques. Elles exigent du temps, de l’engagement et des déplacements sur le terrain qui rendent souvent impossible la présence dans l’hémicycle et en commission. Il est donc légitime d’étendre le champ de ces dérogations aux sénateurs chargés de telles missions. Cet amendement s’inscrit dans une démarche d’équité et de reconnaissance du travail parlementaire sous toutes ses formes. Quel est l’avis de la commission ? Les parlementaires

Nous avons tous ici présidé des assemblées – je le dis à Pierre Ouzoulias, que je remercie de son soutien.

que la parole soit donnée à un seul signataire. Cet amendement vise à préserver la qualité de nos débats, tout en rationalisant nos discussions. En concentrant les interventions, nous gagnons en efficacité sans sacrifier la richesse des échanges. Nous le savons tous, la qualité d’un débat se mesure non pas au nombre d’interventions, mais à leur pertinence. L’objectif n’est bien évidemment pas de restreindre le droit d’amendement, qui est constitutionnel, mais d’éviter les répétitions inutiles qui ralentissent le travail législatif et nuisent parfois à la clarté du débat.

est à M. Michel Masset. La procédure de législation en commission (LEC) a été instaurée pour alléger nos débats en séance publique tout en garantissant un examen approfondi des textes en amont. Cet amendement s’inscrit dans cette logique d’efficacité

Toutefois, nous proposons de fixer la durée de la discussion générale à trente minutes. Il s’agit non pas de remettre en cause le droit des parlementaires à débattre des conventions internationales, mais de rationaliser le débat, dans le souci d’une meilleure organisation de nos travaux.

procédure antidémocratique, mais il s’avère que, depuis la session 2017 2018, les conventions fiscales sont systématiquement adoptées la procédure normale. Il y a bien une discussion générale et un débat sur ces conventions : avis défavorable.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul, ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. » Notre amendement vise donc simplement à mettre en conformité le règlement du Sénat avec la Constitution.

nécessairement donné de délégation de vote. Telle est la raison pour laquelle nous contestons la constitutionnalité de cette procédure.

nationale : « La décision d’appliquer désormais les dispositions constitutionnelles en ce domaine procède du souci de renforcer la crédibilité de notre assemblée, de lui donner toute la place qu’elle occupe dans nos institutions.

L’objectif de l’article 19 est clair : il vise à renforcer la capacité du Sénat à faire entendre sa voix dans le processus de négociation européenne et à améliorer la manière dont le Sénat prend en compte le cadre réglementaire européen lorsqu’il légifère. C’est une nécessité. conduit naturellement à renforcer la commission des affaires européennes, laquelle a été consacrée dans la Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2008. Elle a pour mission d’instruire les textes soumis au Sénat en application des articles 88 4 et 88 6 de la Constitution, d’informer le Sénat sur les autres documents, mais aussi – je le rappelle – de contribuer directement au dialogue politique avec la Commission européenne par le biais des avis politiques, qu’elle est la seule à pouvoir adopter. J’ai entendu les remarques formulées par Éric Kerrouche lors de la discussion générale et je sais que certains s’interrogent sur les rapports entre la commission des affaires européennes et les commissions permanentes. La force de la commission des affaires européennes réside dans sa composition transversale, qui lui permet de bénéficier de l’expertise des collègues appartenant aux différentes commissions, et ce de façon équilibrée. L’article 19 permettra aussi de trouver un équilibre satisfaisant pour l’examen des propositions de résolution européenne (PPRE) déposées par un sénateur. Celles ci ne seront plus examinées automatiquement par la commission des affaires européennes, qui ne sera plus tenue de les étudier dans un délai d’un mois. C’était un souhait de ma part, tout comme la possibilité d’accélérer la procédure d’adoption d’une position du Sénat. Je veux aussi relever que la commission des affaires européennes, qui peut déjà être consultée sur un projet de loi ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national, pourra désormais l’être sur les textes de loi visant à adapter le droit national au droit européen. La parole est à M. Didier Marie, Marie, sur l’article. L’article 19, relatif à la commission des affaires européennes, nous pose question. Nous nous interrogeons sur les intentions et la valeur ajoutée de cet article, qui vise à réécrire le chapitre XX de notre règlement.

la place majeure et grandissante que prenaient les enjeux européens, ainsi que le nombre important de textes européens à traiter et contrôler. Mais cet article met surtout en lumière le rôle des commissions permanentes dans les procédures européennes, notamment une disposition quasiment tombée en désuétude : la préemption des textes européens, au titre de l’article 88 4 de la Constitution, par la commission permanente concernée – une disposition qui n’existe pas à l’Assemblée nationale. Si la réécriture proposée était adoptée, la commission des affaires européennes ne se saisirait que par dérogation,

Elle a acquis de nouveaux droits dans le processus législatif européen et une consécration institutionnelle. Il nous semble indispensable que le règlement du Sénat aille dans le sens d’un renforcement des droits de cette commission. C’est la raison pour laquelle nous proposerons un certain nombre d’amendements

Marie. Il s’agit, par cet amendement, d’affirmer la place de la commission des affaires européennes dans la procédure législative qui la concerne au premier chef. On peut considérer que celle ci est pleinement légitime à exercer systématiquement les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis lorsqu’une PPRE est examinée en séance publique.

que, lorsqu’une PPRE a été adoptée par la commission permanente, tout président de groupe dispose d’un délai de trois jours pour demander son inscription à l’ordre du jour, sous réserve que cette demande soit agréée par la conférence des présidents. Je demande

que cette commission dispose d’une expertise particulière pour suivre les travaux des institutions de l’Union, mais les commissions permanentes sont tout aussi compétentes pour apprécier la dimension européenne des textes dont elles sont saisies

Marie. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité, introduite par la présente proposition de résolution, pour le Gouvernement de demander l’inscription en séance publique d’une proposition de résolution portant avis motivé au titre du principe de subsidiarité.

La procédure concernant les avis motivés au titre de l’article 88 6 de la Constitution vise à ce que ceux ci soient transmis directement au président du Parlement européen, au président du Conseil de l’Union européenne et au président de la Commission européenne, contrairement aux résolutions au titre de l’article 88 4 qui, elles, sont destinées au Gouvernement. Cette possibilité d’inscription en séance accordée au Gouvernement serait, par conséquent, source de confusion et contraire à nos principes.

Il vise à donner à la commission des affaires européennes les mêmes compétences que les commissions saisies pour avis lorsqu’une proposition de résolution portant avis motivé doit être examinée en séance. Mais je connais déjà la réponse de la rapporteure…

par cohérence avec le code de conduite applicable à ces derniers qui leur interdit cette pratique. Entre temps, la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France a introduit un dispositif d’encadrement spécifique des activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger, qui entrera en vigueur au plus tard le 1 juillet prochain. Ce dispositif prévoit des obligations déontologiques renforcées pour les personnes agissant pour le compte d’un mandant étranger, par exemple des cabinets de conseil ou d’affaires publiques, à l’exception des personnels diplomatiques et des agents d’États étrangers agissant dans l’exercice de leurs fonctions, qui ne relèvent pas de cette catégorie. Par cohérence, l’amendement tend à étendre l’interdiction d’accepter des cadeaux de plus de 150 euros aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger. qui pourrait être source d’insécurité juridique pour les sénateurs. L’amendement vise à renvoyer au Bureau du Sénat le soin de définir les invitations à des déplacements qui présentent un lien avec l’exercice du mandat.

de représentant d’intérêts est très large et peut être entendue de diverses manières. Il nous paraît important que le lien avec l’activité parlementaire puisse être apprécié par le comité de déontologie.

constante et ancienne du comité de déontologie a toujours su faire la différence dans les activités que peut englober la notion de déplacement entre ce qui relève du lien avec l’exercice du mandat et ce qui n’en relève pas – je pense, par exemple, à des déplacements de l’ordre de l’agrément personnel, par nature sans lien avec l’exercice du mandat.

et doit rester, celui de la confidentialité de ces décisions

l’enveloppe affectée aux crédits des collaborateurs soit indexée sur l’inflation. Depuis 2020, le salaire moyen des collaborateurs n’a augmenté que de 6

plus professionnelles et donc mieux payées.

de vote. Nous partageons tous la conviction des auteurs des trois amendements quant au fait que la démocratie parlementaire implique, pour son bon fonctionnement, de nous doter des moyens humains nous permettant d’exercer correctement nos mandats. Nos collaborateurs sont des rouages indispensables au bon fonctionnement de l’institution sénatoriale. Ils doivent être en nombre suffisant et rémunérés à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Il me paraît cependant important de rectifier quelques uns des chiffres qui viennent d’être énoncés. Depuis 2018, la rémunération moyenne des collaborateurs a progressé de 12,8 % quand, sur la même période, l’inflation a été de 13,9 %. Le différentiel est donc

Le Sénat n’a pas laissé le pouvoir d’achat des collaborateurs se dégrader sans prendre de mesures correctrices. Depuis l’augmentation de cette enveloppe, intervenue fin 2018, nos collaborateurs ont bénéficié en 2022, puis en 2023, des augmentations du point de la fonction publique, comme les personnels du Sénat. Au total, 7,5 millions d’euros ont été investis depuis 2018 pour l’amélioration des rémunérations de nos collaborateurs. En dehors de ces mesures strictement salariales, nous nous sommes attachés à protéger ces derniers des conséquences de l’inflation. Je citerai, par exemple, l’amélioration de la prise en charge de leurs frais de transport entre domicile et lieu de travail ou le choix que nous avons fait de prendre en charge sur la part employeur les augmentations de cotisations décidées ces dernières années par la mutuelle et la prévoyance.

Par ailleurs, certains dispositifs collectifs particulièrement plébiscités par nos collaborateurs n’existent pas à l’Assemblée nationale, comme le plan d’épargne retraite ou le plan d’épargne d’entreprise. Au total, le Sénat dépense en moyenne 82 000 euros par an et par collaborateur, là où l’Assemblée nationale ne dépense que 59 000 euros. Je mets

conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification. J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Il va être